Monsieur le président,

L'un des arguments pour défendre cette nouvelle stratégie est que la hausse pourra attirer certains étudiants de nationalité chinoise ou indienne, pour qui bien souvent un prix élevé de la scolarité est Vous évoquez,

Je vous remercie,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce 22 janvier marquera l'ouverture de la période de formulation des voeux sur Parcoursup.

Je vous remercie,